d'une part, en métropole après la fermeture du dernier bureau de vote métropolitain et, d'autre part, dans les départements d'outre-mer après la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun de ces départements. Cette disposition est problématique, lorsque le scrutin est organisé dans une circonscription électorale unique qui couvre l'ensemble du territoire national. En effet, lors des élections présidentielle et européenne, les résultats des collectivités ultramarines, qui votent la veille, à l'exception de La Réunion, sont communicables dès le samedi soir, quand bien même le scrutin est organisé le lendemain sur le reste du territoire. Cela est susceptible d'influer sur le scrutin organisé le dimanche. La Commission nationale de contrôle électorale en vue de l'élection présidentielle a ainsi proposé, dans son rapport 2017, de modifier le code électoral sur ce point pour interdire, s'agissant d'un scrutin organisé dans une circonscription nationale, toute communication de de résultats aux médias avant vingt heures, heure de Paris. C'est pourquoi il est proposé de compléter l'article L. 52-2 pour les élections organisées dans une unique circonscription. Pour les autres élections, dont les enjeux sont bien plus locaux, l'influence des résultats ultramarins est moins susceptible d'avoir une influence sur le scrutin métropolitain.

Le code électoral interdit les « affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge Toutefois, cette disposition est l'objet d'interprétations fluctuantes par les commissions départementales de propagande et par les juridictions ; certaines ont en effet une conception très extensive de la notion de « combinaison des trois couleurs Ainsi, une commission de propagande a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte y était écrit en lettres blanches. De même, une autre commission de propagande s'est interrogée pour savoir si la couleur fuchsia pouvait être considérée comme étant du rouge. Lors d'une élection présidentielle, certains ont aussi contesté le fait d'avoir une cravate tirant sur le rouge avec un costume bleu marine et une chemise blanche. Récemment, un slogan écrit en bleu en haut d'une profession de foi et suivi par un texte, où les sous-titres étaient soulignés en rouge, a même été contesté. Le rapport établi par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012 livre un intéressant aperçu de cette casuistique casuistique : « S'agissant d'un candidat, la commission a été conduite à refuser d'homologuer ses premiers projets en raison de la proximité du bleu du tissu de la chemise du candidat, du blanc des lettres composant son nom et du rouge des lettres indiquant son site internet ou de la teinte du bas de l'affiche qu'elle a jugée être non pas orange mais rouge sur les exemplaires imprimés sur papier. Sur ces projets, le rapprochement de la teinte rouge avec les lettres blanches du nom du candidat et le tissu bleu apparaissant sur la photographie traduisait, aux yeux de la commission, une combinaison des trois couleurs nationales prohibée par l'article R. 27 du code électoral. En revanche, la commission a estimé que la couleur orange utilisée pour d'autres affiches était bien orange, que le costume d'un candidat s'inscrivait dans la gamme chromatique des noirs et non des bleus, que le point rouge constitué par une décoration nationale épinglée sur le costume d'un candidat ne conduisait pas à voir une méconnaissance de la prohibition d'emploi des trois couleurs nationales faite par l'article R. 27 du code électoral ». En fait, l'interdiction d'utiliser les trois couleurs a pour but d'éviter qu'un document électoral entraîne une confusion avec l'emblème national ou ait indûment un aspect officiel. L'interdiction doit donc être appliquée ... Merci ! ... en tenant compte de ce que la simple présence

j'ai moi-même eu une expérience qui ressemble beaucoup à celle de notre collègue Roger Karoutchi. Je possède une très jolie cravate : elle est rouge, avec des rayures bleues et des canards ... beiges. Je la porte en chaque grande occasion. Aussi, pour me porter chance, la portais-je lors de la photographie qui allait servir à constituer mes documents électoraux. j'ai été extraordinairement vexé que la commission de propagande, qui siège à Villedieu-les-Poêles dans le département de la Manche et qui était présidée par une jeune magistrate, confonde le beige des canards avec du blanc sale.

et qui a l'habitude des documents électoraux, a su lui aussi, ce qui m'a émerveillé, modifier la couleur de ma cravate. À la suite de cette opération, la photographie de mon document électoral était beaucoup moins jolie

Certains ici pensent qu'elle aurait laissé passer ma cravate, d'autres diront le contraire ; quant à la magistrate, je ne sais pas ce qu'elle aurait décidé. Dès lors, si M. Masson a bien fait de poser le problème, je crois que la solution qu'il apporte

l'avis de la commission ? L'amendement n° 15 vise à consacrer l'existence d'un service public national de l'envoi des documents de propagande, donc à interdire à l'État de sous-traiter cette prestation.

comment créer un service public national de ce type ? On imagine mal les agents de l'État distribuer eux-mêmes ces documents de propagande. Ensuite, comment limiter dans la loi la liberté contractuelle de l'État ? Cela nous semble poser un problème de constitutionnalité.

en souhaitant que ces quelques défaillances isolées ne se reproduisent pas et en s'en remettant à la vigilance des services de l'État et, singulièrement, aux consignes qui pourraient être données pour les prochains scrutins par le Gouvernement.

des modalités d'acheminement, de la sous-traitance et du mode de gestion de ce service public. Je rappelle en outre que les préfectures ont fait l'objet d'un plan de modernisation important, qu'elles se sont recentrées sur leurs missions prioritaires et que les personnels sont

Le Conseil constitutionnel n'a pas fait droit aux griefs en cause, dans la mesure où les faits dénoncés, qui n'étaient pas toujours établis, n'avaient pas pu, eu égard aux écarts de voix entre les candidats, avoir d'incidence sur les résultats des scrutins contestés. Toutefois, il a appelé à sécuriser davantage les opérations de mise sous pli et d'acheminement des documents électoraux et à veiller à informer les électeurs en cas de dysfonctionnements. Néanmoins, certains candidats ont livré l'ensemble des circulaires et bulletins de vote et ont été privés de leur acheminement aux électeurs. Ils ont engagé des sommes importantes, dont le remboursement n'est attribué que s'ils ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Je vous propose donc que les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés soient également remboursés de leurs frais engagés en cas de défaillance avérée

remarquable, avec la mise sous pli. Monsieur Grand, il ne nous semble pas que la réponse aux difficultés réelles que vous évoquez soit de rembourser les candidats qui n'ont pas atteint le seuil de suffrages imposé par le législateur pour bénéficier de la prise en charge des dépenses électorales. électorales. Une défaillance logistique ne doit pas donner un droit supérieur à celui qui est acquis par l'élection ni invalider une décision souveraine de la Commission nationale des comptes de campagne

lors des dernières élections européennes. Nous comprenons parfaitement votre préoccupation, mais je rejoins la remarque de M. le rapporteur sur la nécessité de veiller à ce que les routeurs exécutent correctement leur mission et à l'application ferme et stricte des sanctions financières. L'avis est défavorable. La parole est

la défaillance des routeurs et que, s'ils ne font pas leur travail, ils seront sanctionnés. Je serais tenté de dire que ce n'est pas non plus au candidat de payer la défaillance de l'État et des routeurs. Je retire mon amendement, mais je vous demande quand même de vous pencher sur la question. Pour dix voix,

Le problème, ce n'est pas de faire payer le routeur qui n'a pas fait son travail ou de rémunérer les postiers. Le vrai problème, c'est le candidat qui est spolié,

Mes chers collègues, Il est pertinent d'interdire la reproduction de photographie de personnes sur le bulletin de vote. En revanche, nul ne sait à l'avance quel sera le candidat qui devra ensuite présider l'organe délibérant concerné par le scrutin. La disposition correspondante de la proposition de loi crée donc la confusion. Par exemple, dans le cas d'une élection législative, nul ne peut dire à l'avance qui sera candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. La proposition de loi pourrait donc conduire à des dérives et à des abus, car on ne peut pas empêcher un candidat de prétendre que telle ou telle personnalité a vocation à être président de l'Assemblée nationale. Il en est également de même pour les élections locales, car, bien souvent, à l'issue du premier tour, les tractations politiques conduisent à des accords très différents de ce qui était initialement prévu. Quel est l'avis de la

conseillère municipale sur cette liste, une fois que je serai élue conseillère départementale au scrutin uninominal, je voterai pour telle ou telle personne pour la présidence de l'exécutif. Je ne vois pas en quoi il y a malice, remise en cause de la démocratie ... Merci ! ... ou défiance à l'égard de nos électeurs. Louis Masson, pour explication de vote.

la personne qui a vocation à être candidate à la présidence ? Si vous avez 1 000 candidats à une élection départementale, il y a 1 000 personnes qui ont vocation à être candidates à la présidence

parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote. Plus rien ne va ... J'envisageais, sur mon prochain bulletin de campagne sénatoriale, de mettre les photos de Macron et de Sarkozy, et je vois qu'on veut tout m'interdire.

Quand on instaure une interdiction, il faut toujours le faire avec mesure et réflexion, dans un domaine qui est, par définition, celui de la liberté et du pluralisme

j'ai le plaisir de saluer, dans la tribune d'honneur du Sénat, une délégation de six députés du groupe d'amitié Égypte-France de la Chambre des représentants de l'Égypte, conduite par le Dr Ayman Aboul Ela. Ils sont accompagnés par notre collègue Mme Catherine Morin-Desailly, présidente du groupe interparlementaire d'amitié France Égypte. La délégation est en France jusqu'au 29 juin pour une visite d'étude consacrée notamment au développement de nos coopérations économiques, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables et des transports. La délégation s'est rendue lundi dans les Yvelines pour visiter le site de la société Colas, filiale de Bouygues, afin d'étudier le projet de la route solaire Wattway, en cours d'expérimentation sur plusieurs sites en France et à l'étranger. Elle se rendra en fin de semaine à Toulouse pour visiter le site d'Airbus. Le Sénat français entretient d'excellentes relations de confiance et d'amitié avec le Parlement égyptien, relations qui ont vocation à s'intensifier à la suite du référendum d'avril, par lequel le peuple égyptien s'est prononcé, notamment, en faveur de la création d'un Sénat, lequel avait été temporairement supprimé. Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter, en votre nom à tous, à nos homologues du Parlement égyptien, la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'un excellent et fructueux séjour.

une petite anecdote. En 1965, Louis Pradel s'est présenté à la mairie de Lyon. À l'époque, il n'était pas possible de faire figurer son nom dans l'ensemble des arrondissements.

un choix de premier tour et, ensuite, il y a des ralliements et des fusions pour le second tour, avec des alliances possibles. Ça ne me choque donc pas que des gens qui ont rêvé

les noms, participe aussi au lien de proximité entre les citoyens et leurs représentants. Cet amendement vise donc à maintenir la possibilité de faire figurer la photo du candidat ou de son remplaçant sur le bulletin de vote. Quel est l'avis de

et noble de retenir le nom, le symbole politique ou le sigle politique de tel ou tel, alors qu'il serait bassement populaire et antidémocratique de retenir la photographie ou le visage de telle personne qu'on a rencontrée au cours d'une campagne électorale ?

Comme vous le savez, le code électoral prévoit que pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors des emplacements spéciaux réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. Outre une violation du code électoral, l'affichage électoral sauvage constitue également une pollution sanctionnée par le code de l'environnement, et le maire peut saisir le préfet en vue de prononcer une amende forfaitaire prévue par ce même code. Or ces dispositions ne suffisent pas pour lutter contre la prolifération de l'affichage électoral sauvage.

s'inspirant de la jurisprudence du tribunal administratif de Grenoble, il est proposé, par cet amendement, que le coût induit par le nettoyage incombe au candidat que l'affiche promeut et que le maire puisse procéder à la dépose d'office des affiches après une mise en demeure restée vaine. Pour ne pas créer une nouvelle sanction administrative que certaines autorités municipales ont déjà des difficultés à faire respecter, il est simplement suggéré de reporter ce coût sur les remboursements des dépenses de propagande électorale, sauf apport sauf apport de la preuve par les candidats en cause qu'ils ne sont pas à l'origine de cet affichage illicite. Quel

Il se trouve que cette infraction d'affichage sauvage fait déjà l'objet de six sanctions : la voie civile, le juge des référés peut contraindre le candidat à enlever ses affiches ; la voie pénale, l'affichage sauvage est puni de 9 000 euros d'amende la voie administrative, le maire peut ordonner la dépose des affiches et le remboursement des frais exposés par le candidat ; la voie environnementale, avec une amende de 1 500 euros, sans compter la perception par les électeurs de la pollution la voie électorale, le juge annulant le scrutin lorsque les affiches ont trompé les électeurs. En outre, il est vrai- je rejoins notre collègue Reichardt -qu'il existe une dernière voie, souvent méconnue lorsque l'affiche remplit certaines conditions, le maire ou le préfet peut demander au candidat de la déposer et de mettre les lieux en état dans un délai de deux jours. L'amendement vise à aller un petit peu plus loin, en explicitant la possibilité pour le maire de déposer d'office les affiches électorales- la jurisprudence le permet déjà -, mais il prévoit aussi que le coût du nettoyage serait imputé sur le remboursement des dépenses électorales des candidats, avec les risques induits d'inéligibilité et la création d'une nouvelle sanction.

de lutte contre l'affichage sauvage, il nous faudrait travailler plus en profondeur sur l'articulation entre les dispositifs déjà existants et sans doute sensibiliser les maires-

Gouvernement ? Comme vient de le préciser M. le rapporteur, il existe plusieurs dispositions légales qui viennent d'ores et déjà sanctionner cet affichage sauvage. Je rappelle que la proposition de loi que nous examinons vise à clarifier certaines dispositions du code électoral. Les dispositifs concernant l'affichage sauvage sont sans doute

La parole est à M. Jean-Pierre Grand. L'article 5 insère dans la partie législative du code électoral des dispositions contenues dans sa partie réglementaire. Il s'agit de rappeler l'interdiction de faire figurer sur le bulletin de vote d'autres noms de personne que celui des candidats. On va rouvrir le débat Pour les scrutins de liste, cette règle est fréquemment détournée par l'insertion du nom d'une ou de personnes non candidates dans le titre de la liste. Ainsi, lors des élections régionales de 2015, les listes du Front national s'intitulaient « Liste Front national présentée par Marine Le Pen », quand, dans un même temps, celle-ci menait dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie une liste intitulée « Une région fière et enracinée ». Or le titre de la liste doit figurer obligatoirement sur le bulletin de vote. Afin de rendre réellement effective cette interdiction, je vous propose d'interdire également l'utilisation dans le titre de la liste, choisi lors de la déclaration de candidature, d'autres noms de personne que celui des candidats. Lors de l'examen en commission, le rapporteur a précisé que cet amendement était partiellement satisfait par l'article 5. Mais il convient d'aller au bout de la logique de cette interdiction.

Gouvernement ? Les titres des listes doivent rester un espace de liberté. Autant il paraît justifié de renforcer la réglementation des bulletins de vote, car ces derniers peuvent induire en erreur l'électeur le jour du vote quand la propagande n'est autant le libellé de la liste relève du contenu de la campagne électorale dont il semble difficile de limiter le contenu. Pour l'ensemble est ainsi libellé : La parole est à M. Jean-Pierre Grand. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les bulletins de vote doivent comporter au regard du nom des candidats ressortissants des États membres de l'Union européenne autre que la France l'indication de leur nationalité. Face à l'augmentation du nombre de contentieux, je vous propose de prévoir le non-remboursement des frais d'impression des bulletins de vote pour les listes de candidats aux élections municipales n'ayant pas respecté cette règle. prévoir une sanction financière en parallèle de la proposition de suppression de la nullité de l'élection en cas de non-respect de cette obligation, que je défendrai lors de l'examen de la proposition de loi organique.

s'agissant de l'encadrement des élections sénatoriales, sont liées non à la volonté du législateur mais à une absence de renvoi dans le code électoral. Cet apport de la commission, qui réinscrit l'élection sénatoriale

La loi du 11 décembre 1990 visait les modifications effectuées par décret, à savoir, pour l'essentiel, le redécoupage des cantons. Certaines personnes prétendent même que ce pseudo-usage républicain

comme l'indique l'exposé des motifs de la loi du 11 décembre 1990, c'est une sorte de fossile législatif, qui doit être abrogé. Pour le reste, il n'y a aucune raison de consacrer un « usage républicain » qui n'a rien de républicain et qui n'existe pas ! L'argument souvent évoqué selon lequel il n'est pas possible de modifier les règles électorales moins d'un an avant un scrutin est faux. En mars 2014, les élections municipales se sont déroulées sur la base de la loi du 17 mars 2013, laquelle avait considérablement modifié le mode de scrutin. De même, en 2008, pour les élections cantonales, la loi avait été modifiée à peine un mois avant le scrutin, et cela déjà pour des questions de parité, alors même que les opérations préparatoires au scrutin avaient déjà débuté.

par ses : « Les sénateurs invoquaient, en premier lieu, la tradition républicaine qui veut qu'on ne procède pas à une modification des règles électorales dans l'année qui précède un scrutin et,, lorsque le processus électoral a débuté. Le grief avait été soulevé au cours des débats. L'opposition avait d'ailleurs déposé, en vain, dans les deux assemblées, un amendement tendant à reporter l'entrée en vigueur de la loi au 1 janvier 2009. Il est vrai que ce délai d'un an a été le plus souvent respecté. Mais il ne l'a pas toujours été et n'a jamais été consacré par aucune loi de la République ; il ne pouvait donc se voir reconnaître la valeur d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme le demandaient les requérants. » Quel est l'avis de la ? Mme Kauffmann vient de faire la démonstration que cette tradition républicaine n'est pas toujours respectée. Précisément, les dispositions qu'elle nous demande de supprimer visent à inscrire dans la loi

notre amendement n° 26 : il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la présente loi aux prochaines élections municipales, notamment pour ce qui concerne la présentation des bulletins de vote.

n° 26 : il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la présente loi aux prochaines élections municipales, notamment pour ce qui concerne la présentation des bulletins de vote.

L'instauration du quinquennat et la fixation de la date des élections législatives juste après l'élection présidentielle ont, d'une certaine manière, dévalorisé les élections législatives aux yeux des Français. Nombre d'entre eux ont le sentiment que l'enjeu principal est déjà tranché et que l'élection des députés n'est plus que la confirmation du choix opéré pour le Président de la République. Il existe un moyen simple d'enrayer cette dérive : organiser en même temps l'élection du Président de la République et celle des députés. Une telle mesure contribuerait également à réduire l'abstention lors des élections Enfin, cette simultanéité des deux scrutins favoriserait le pluralisme. Les électeurs qui, au premier tour de l'élection présidentielle, ont exprimé leur préférence pour un candidat ayant peu de chances de figurer au second tour voteraient en effet plus volontiers pour sa formation politique aux élections législatives si celles-ci avaient lieu en même temps. Une telle réforme implique de compléter l'article L.O. 122 du code électoral. Bien entendu, les dispositions en cause n'auraient pas lieu de s'appliquer en cas de décès ou de démission du Président de la République, ou en cas de dissolution de l'Assemblée nationale.

obligera peut-être le juge à prouver la volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité en toutes circonstances, alors que, à l'heure actuelle, il ne peut apporter cette preuve dans deux cas sur trois, parmi ceux qui sont énumérés. Par ailleurs, la constance de la jurisprudence montre que les erreurs matérielles ne donnent pas lieu à une inéligibilité et que le juge peut mettre en oeuvre une proportionnalité de sanctions. Cette différence de lecture fondamentale

En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales par le candidat, ou si celui-ci n'a pas déposé son compte de campagne, le juge peut prononcer

du nom de ces candidats l'indication de leur nationalité. L'absence de cette précision entraîne la nullité du bulletin de vote et, bien souvent, l'annulation des élections. Dans les faits, on distingue deux situations. Soit les bulletins sont pris en compte dans le dépouillement, auquel cas il reviendra au juge administratif de réviser le résultat de l'élection, ou de l'annuler, en fonction des suffrages obtenus par la liste en cause et des conséquences sur la sincérité du scrutin. les bulletins sont considérés comme nuls lors du dépouillement, auquel cas il reviendra au juge administratif de se prononcer sur l'impact de cette non-comptabilisation sur la sincérité du scrutin. Le juge administratif prend ces décisions en fonction du nombre de voix obtenu par la liste ; il mesure l'impact sur le résultat du poids des électeurs qui n'ont pas été en mesure d'exprimer valablement leur suffrage. Afin de sécuriser les opérations de vote, il est donc proposé de supprimer ce motif de nullité au regard de la faible importance de cet oubli de pure forme. J'en reviens à ce que je disais : ne laissons pas les jurisprudences faire la loi ! Les candidats doivent préciser leur nationalité sur le bulletin de vote, à peine de nullité. M. Grand souhaite revenir sur ce motif de nullité et comptabiliser les bulletins en questions.

qu'une telle mention était nécessaire à l'information des électeurs, dès lors que les conseillers municipaux n'ayant pas la nationalité française ne peuvent ni exercer des fonctions communales exécutives ni participer à l'élection des sénateurs. Par suite, cette mention ne revêt pas de caractère discriminatoire. Dans cette même décision, et par le Conseil constitutionnel avait jugé que l'indication de la nationalité des ressortissants de l'Union européenne candidats dans des communes de 2 500 habitants et plus, prévue à peine de nullité par code électoral, n'était pas contraire au principe de non-discrimination. Dès lors, loin de constituer une complication administrative superflue, cette règle traduit concrètement une obligation de nature constitutionnelle, qui impose d'annuler les bulletins de vote ne comportant pas cette mention. Le Gouvernement émet donc

La loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a créé un nouveau mécanisme d'inéligibilité pour les parlementaires qui ne respectent pas leurs obligations fiscales.

Comme l'a indiqué le Gouvernement au cours de nos auditions, il est important de sécuriser l'inéligibilité prononcée pour un manquement aux obligations fiscales. Il s'agit, tout simplement, de confirmer que, si les parlementaires concernés ont l'interdiction, pendant la durée de leur inéligibilité, de se présenter à d'autres scrutins,

d'une reprise de la disposition qui figure aux articles L.O. 136-1 et L. 136-3, qui prévoient respectivement des sanctions d'inéligibilité dans le cas d'un dépassement du plafond de dépenses électorales et de manoeuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin. Cette précision ne remet donc absolument pas en cause la compétence du Conseil constitutionnel pour prononcer l'inéligibilité ainsi que la démission d'office d'un député, comme il l'a fait dans sa décision du 6 juillet 2018. Elle rend simplement explicite l'absence de conséquence sur les mandats acquis antérieurement, comme cela avait d'ailleurs été le cas à la suite de la décision mentionnée. Le Gouvernement

Le scrutin est ouvert.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre des réseaux radioélectriques mobiles

vous examinez aujourd'hui en première lecture en séance publique la proposition de loi sur le déploiement de la 5G et la sécurité de nos réseaux. Cette lecture est éclairée par le rapport de Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires économiques.

les États qui sauront en massifier l'usage sont susceptibles de prendre une avance technologique, notamment en matière industrielle. Il faut donc se donner les moyens non seulement de déployer la 5G en France, mais surtout d'en développer les usages, tant industriels que de services, pour renforcer notre compétitivité.

c'est-à-dire à la création de plateformes d'expérimentations où n'importe quelle entreprise, fût-elle une PME ou une entreprise de taille intermédiaire, peut venir tester son produit Les modalités sont simples : pendant trois ans, ces plateformes seront autorisées à utiliser des fréquences 26 gigahertz, et les innovations pourront être testées en s'affranchissant en partie du cadre réglementaire. France est, semble-t-il, avec l'Allemagne, la plus avancée dans cette démarche. C'est un levier pour gagner du terrain et acquérir une avance technologique. La troisième orientation consiste à préserver la sécurité de nos réseaux et de nos communications. Tel est l'objectif du texte qui vous est aujourd'hui Dans cette perspective, tous les équipementiers sans distinction doivent être soumis aux mêmes règles, car des vulnérabilités ou des failles de sécurité peuvent être constatées chez tous les équipementiers. En outre, les actionnariats et les stratégies des équipementiers peuvent évoluer dans le temps. Quand on parle de 5G, je le rappelle, on parle de temps long- dix à quinze ans au minimum. À ce titre, il convient d'être très vigilant. Finalement, cette nouvelle protection ne doit pas retarder l'innovation et la réussite de la 5G. Il me semblait nécessaire de rappeler ces grands principes

je ne partage pas la critique que vous nous avez adressée d'avoir voulu « passer en force ». Depuis nos premiers échanges dans le cadre de l'examen du projet de loi Pacte, nous avons eu de longs débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nos débats en commission, dans cette assemblée, ont permis de simplifier et de clarifier le dispositif. Je pense à la précision sur le champ d'application du dispositif pour le limiter aux équipements de cinquième génération et de générations ultérieures. Nous écoutons, nous débattons et nous améliorons le texte. Madame le rapporteur, vous avez également émis des propositions. la commission a supprimé la mention du périmètre géographique d'exploitation dans le dossier de demande. Comme je l'ai affirmé lors de mon audition en commission, il n'est pas question que l'État dicte aux opérateurs leur politique d'achat. Le Gouvernement est donc favorable à cette proposition de clarification, qui est particulièrement bienvenue. La proposition d'instaurer une autorisation du Premier ministre sous condition me semble en revanche présenter des risques contentieux. La sensibilité du Sénat sur les questions de couverture numérique du territoire est tout à fait compréhensible, et le nouveau dispositif doit être conçu pour avoir un minimum d'impact sur les déploiements des opérateurs. Le fait de qualifier des décisions de deux mois

également poser un problème au regard du principe de la liberté d'établissement au sein de l'Union européenne, d'autant plus que l'effort de protection de la sécurité des futurs réseaux 5G se déroule dans le cadre d'une démarche coordonnée à l'échelon de l'Union européenne, au sein de laquelle la France entend pleinement prendre sa part en partageant des informations avec ses partenaires.

dans la gestion des réseaux français ; cela ne serait pas possible au regard du droit européen. Le Gouvernement souhaite donc revenir à la version du texte voté par l'Assemblée nationale, car il considère que cette évolution

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, on pourrait décrire la 5G comme la génération des superlatifs. Elle nous promet des débits multipliés par dix, un temps de latence divisé par dix, des réseaux plus flexibles, plus fiables, moins énergivores Elle permettrait, grâce à ses nouvelles caractéristiques, le développement de nouveaux usages, tels que l'usine ou la maison connectée, ou encore le véhicule du futur. S'il convient de garder une certaine distance par rapport aux promesses commerciales, il faut cependant prendre au sérieux les apports de cette technologie à l'économie d'un pays, comme en atteste la véritable course à la 5G qui s'est engagée, sur tous les continents, en vue de bénéficier en premier de ses retombées économiques. Le Gouvernement entend y prendre sa part, grâce à la mise en oeuvre de sa feuille de route sur la 5G. la criticité des usages nécessite également de rehausser le niveau d'exigence quant à la sécurité de ces réseaux. C'est l'objet de la « proposition de loi »- j'utilise les guillemets En instaurant un régime d'autorisation préalable à l'exploitation de certains équipements des réseaux 5G, ce texte entend conférer au Premier ministre le moyen de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Le Gouvernement estime, en effet, qu'une évaluation de la sécurité des réseaux de bout en bout s'impose avec la 5G, contrairement aux générations précédentes où une approche centrée sur l'analyse des équipements suffisait. L'affaire Snowden a montré la vulnérabilité des réseaux de télécommunications. Avec la 5G, l'espionnage, l'altération des messages, l'indisponibilité du réseau ou une attaque informatique massive pourraient avoir des conséquences catastrophiques pour un pays. Il convient donc d'anticiper le plus en amont possible, en rehaussant le niveau de sécurité exigé. Nombreux sont les pays qui réfléchissent à cette question. Certains pensent avoir trouvé la solution en interdisant l'équipementier chinois. C'est le cas des États-Unis, ce n'est pas l'orientation du Gouvernement, vous l'avez confirmé, madame la secrétaire d'État, ni celle du Sénat- et c'est heureux. Certes, notre pays n'a pas tout à fait la même conception de la liberté que la Chine, mais, j'insiste, nous ne sommes pas non plus à l'abri d'une nouvelle affaire Snowden, déploiement de la 5G, aurait des conséquences bien plus dramatiques ! Nous partageons donc avec le Gouvernement le même constat : une élévation du niveau des exigences de sécurité sur la 5G est nécessaire. Nous avons tous à y gagner quel serait l'intérêt de recourir à un réseau dans lequel nous n'avons pas confiance ? Je crois que nous pourrons aussi être d'accord sur l'intérêt du bicamérisme et des débats parlementaires nourris

Madame la secrétaire d'État, si vous n'en étiez pas encore convaincue, je crois que nous faisons ainsi la démonstration que le bicamérisme et les débats parlementaires permettent de clarifier les choses et d'améliorer les textes Qu'a voulu faire la commission des affaires économiques ? Tout simplement éviter que le Gouvernement ne dévie de la trajectoire qu'il s'est fixée dans sa feuille de route sur la 5G, et cela en tentant de trouver un équilibre juste entre les impératifs de sécurité et les besoins des entreprises et des usagers de la 5G. Je souligne d'ailleurs que, si le Gouvernement a publié sa stratégie sur la 5G deux ans après la Commission européenne, il est cependant pionnier sur la question de la sécurité, en proposant une initiative législative quelques mois avant que la Commission Les esprits taquins pourraient être tentés de dire que notre pays est toujours en retard quand il s'agit d'accompagner l'innovation, mais toujours en avance quand il s'agit de la brider ou de légiférer Fort heureusement, ce n'est pas le cas de la commission des affaires économiques, qui a modestement souhaité maintenir le cap de la sécurité tout en répondant aux inquiétudes nombreuses que ce texte a pu faire naître : celles de nos concitoyens, qui en ont assez d'être laissés au bord du chemin numérique ; celles de nos entreprises, ensuite, qui entendent accéder aux réseaux pour innover, quel que soit leur lieu d'implantation ; celles des opérateurs, enfin, qui ne veulent pas qu'on leur impose de construire des réseaux militaires à la place des réseaux civils. Nous avons donc fait en sorte que le texte soit davantage proportionné. Nous l'avons également précisé et simplifié. Ainsi, nous souhaitons nous assurer que l'approche du Premier ministre sera proportionnée aux risques. Nous avons entendu vos propos sur ce sujet, madame la secrétaire d'État, et je ne doute pas que le Premier ministre connaisse le sujet sur le bout des doigts, mais, si les hommes et les gouvernements

Nous avons aussi précisé que le texte ne s'appliquerait qu'aux équipements des réseaux 5G, inscrivant ainsi dans le marbre l'intention du Gouvernement, afin de limiter les effets de bord sur les déploiements de la 4G qui sont en cours. Je pense que cette disposition rassurera bon nombre de mes collègues. Afin d'éviter de recréer un ministère des PTT qui dicterait aux opérateurs, sous la haute autorité du Premier ministre, leur politique d'achat, nous avons également supprimé la mention du périmètre géographique dans le dossier de demande. Madame la secrétaire d'État, nous avons apprécié que vous nous suiviez sur ce point. économiques a également entendu éviter de créer des surcharges administratives en fusionnant le régime applicable aux opérateurs dans le cadre de l'article R. 226-7 du code pénal avec celui de la présente proposition de loi.

Je tiens enfin à saluer le travail du rapporteur pour avis, Pascal Allizard. Nous avons travaillé en bonne intelligence, comme le montre l'adoption, par notre commission, des améliorations qui nous ont été proposées par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Fidèle à la démarche que j'ai adoptée depuis le début sur ce texte, je souhaite que nos débats soient constructifs et nous permettent d'envisager une commission mixte paritaire dans l'intérêt de tous, en particulier celui de la France et de sa compétitivité.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, madame le rapporteur mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné la proposition de loi le 12 juin dernier et donné un avis favorable à son adoption. Elle estime important et urgent de prendre des dispositions législatives pour assurer une meilleure résilience des réseaux de télécommunications, dont la criticité est déjà élevée et va s'accroître, car ils seront le support du développement exponentiel de services essentiels à la vie économique et à la vie quotidienne de nos concitoyens. La fiabilité des réseaux, leur protection contre des attaques informatiques à des fins d'espionnage, de déni d'accès, mais aussi de sabotage, doit être maximale et leur résilience à la hauteur de leur vulnérabilité. Compte tenu des enjeux, certaines interruptions de service pourraient causer des dommages aussi importants que certaines catastrophes naturelles. Il est donc légitime que la protection des intérêts de la défense et de la sécurité nationale soit prise en considération avant leur déploiement. La commission des affaires étrangères et de la défense a souscrit à ce texte pour cinq raisons. Premièrement, ce régime est nécessaire. Les régimes actuels relevant soit de la protection de la correspondance privée, soit de la protection des systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale, sont inadaptés et insuffisants. Deuxièmement, ces règles sont adaptées à l'évolution technologique majeure des réseaux apportés par la 5G, à savoir la redistribution de l'intelligence des équipements, du coeur de réseau vers les stations de base des antennes, à sa périphérie, et la virtualisation croissante de leurs composantes, qui reposeront davantage sur des logiciels. Troisièmement, le régime proposé est fondé sur la responsabilité des opérateurs, qui doivent être en mesure de garantir de bout en bout la sécurité de leurs réseaux et d'assurer la puissance publique de la fiabilité des matériels et logiciels installés, de la qualité de l'organisation mise en oeuvre et de leurs fournisseurs et sous-traitants.

Il permet de prendre en compte, si nécessaire, le risque qui pourrait résulter « du fait que l'opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitante, soient placés sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'une puissance étrangère », et ce sans créer d'interdit général et absolu à l'encontre d'aucun.

et qui s'est montrée attentive à nos observations. Là aussi, je l'en remercie. La commission des affaires étrangères a également pris soin de vérifier, à défaut d'étude d'impact, que les moyens en personnel dont disposera l'Anssi pour instruire ces demandes ont bien été anticipés dans la montée en puissance de cette agence agence dans le triennal budgétaire. La commission des affaires étrangères considère aussi que ce régime devra faire l'objet d'une évaluation au regard de l'évolution des usages et du développement des technologies,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la France est parmi les premiers pays à se doter d'un cadre visant à préserver ses intérêts économiques et politiques en matière de réseaux radioélectriques mobiles. Par ce texte, elle instaure une nouvelle autorisation préalable à l'exploitation des équipements de réseaux, venant étendre le champ de l'article R. 226-3 du code pénal, qui prévoit déjà une autorisation à la commercialisation et à la détention d'équipements de réseau pouvant porter atteinte au secret des correspondances électroniques.

nationale. Avec la 5G, les risques en matière de cybersécurité et de souveraineté nationale sont accrus. Ils sont liés aux équipements du réseau et à ses spécificités techniques, notamment sa plus grande surface de vulnérabilité à d'éventuelles attaques, mais également au champ très vaste de ses usages touchant des activités sensibles. Il est donc essentiel de se prémunir contre des risques de piratages, d'attaques, d'espionnage ou simplement d'indisponibilité, qui pourraient engager la vie de personnes. La difficulté de l'exercice vient de ce que ces risques ne sont pas encore bien identifiés et qu'ils sont de nature à évoluer. Les équipementiers, les opérateurs, les fabricants de smartphones et de terminaux comme les éditeurs de contenus et de services sont tous touchés par cet enjeu de sécurité qu'ils ont eux-mêmes qualifié d'holistique. Ils ont souligné que « la diversité des équipementiers constitu[ait] également un gage de sécurité Parallèlement à cet impératif de sécurité, l'État doit progresser rapidement dans l'attribution des fréquences 5G, pour préserver la compétitivité des entreprises françaises. Il doit dans le même temps veiller ce que ces nouvelles obligations ne viennent pas perturber le déploiement actuel de la 4G. La proposition de loi que nous examinons vise à instaurer ce nouveau cadre réglementaire sur la sécurité et l'intégrité des réseaux de télécommunications, avant même l'arrivée de la 5G. Mme le Mme le rapporteur Catherine Procaccia a souhaité procéder à un rééquilibrage de ce texte, entre exigence de protection des libertés économiques et approche sécuritaire. Je salue son travail sur ce sujet complexe et évolutif. Elle a orienté ses propositions autour de trois axes opérationnels et proportionnels : rééquilibrer, simplifier et préciser. Dans cette phase de cadrage du dispositif, je tiens à souligner le rôle décisif de contrôle et de veille

Il nous semble également important d'appréhender les périmètres géographiques lors des déploiements. Ils ont, à juste titre, été supprimés de la demande d'autorisation pour des motifs économiques. Néanmoins, il convient qu'ils soient portés à la connaissance de l'administration en charge de la sécurité des équipements sensibles. Nous l'avons dit lors de l'examen de ce texte en commission, nous ne sommes qu'au début d'une régulation qui devra s'adapter aux pratiques et aux progrès technologiques. En ce sens, nous serions favorables à la remise d'un rapport annuel au Parlement et à la formation d'un groupe de suivi 5G, permettant aux parlementaires de s'assurer de la pertinence des dispositions en vigueur. La 5G est le relais de croissance, le moteur de l'économie de demain. L'enjeu de son déploiement rapide est fondamental. En conséquence et moyennant les précisions évoquées, le groupe Union Centriste soutiendra ce texte.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, l'actualité récente a fait naître un climat de défiance, mais aussi une prise de conscience des enjeux liés à la sécurité des réseaux 5G. Un équipementier majeur a été montré du doigt et accusé d'espionner ses clients. Face à ceux qui crient au loup, nous nous réjouissons que la France choisisse de répondre avec sang-froid, mais sans naïveté. L'objet de la proposition de loi que nous examinons cet après-midi est de proposer un cadre sécuritaire pour le développement de cette technologie. Les réseaux radioélectriques mobiles sont à l'aube d'une transformation fondamentale, si fondamentale qu'il nous est difficile d'en prévoir les évolutions et de savoir la technologie 5G est porteuse de risques, parce qu'elle est nouvelle, parce que son architecture est très différente de celle de la 4G, parce que les usages auxquels elle est destinée sont eux-mêmes sensibles, parce qu'elle consacrera l'internet des objets, multipliant ainsi les accès au réseau et, par là même, les failles potentielles. Malgré ces risques, la France a tout de même choisi de franchir ce cap. Nous nous en réjouissons, car les possibilités offertes par cette technologie sont monumentales. Il nous appartient de définir les modalités de son usage, afin qu'il se réalise dans les meilleures conditions. L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique », affirmait Albert Einstein. Nous ferions bien de nous en souvenir. Le groupe Les Indépendants se félicite toujours de l'initiative parlementaire. Il est toutefois plus réservé lorsque la complexité d'un sujet rend particulièrement éclairantes, sinon nécessaires, la réalisation d'une étude d'impact et la saisine du Conseil d'État pour avis qui accompagnent les textes. Cette proposition de loi aurait ainsi pu grandement bénéficier de tels éclairages. Au-delà de ces considérations, nous estimons que le dispositif envisagé est pertinent. En particulier, il nous semble de bonne économie de faire peser la demande d'autorisation sur les opérateurs télécoms désignés comme « opérateurs d'importance vitale Plusieurs options étaient possibles, mais celle-ci nous paraît servir le mieux l'objectif de sécurité nationale, à savoir s'assurer que les réseaux télécoms soient opérationnels et fiables, quel que soit l'équipementier choisi. Nous avons toute confiance dans la compétence des services du Premier ministre, au premier rang desquels le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, pour mener à bien l'examen préalable à l'autorisation d'exploitation. Nous sommes également satisfaits par l'approche de ce texte, qui a vocation à s'appliquer à tous sans discrimination. C'est juste, car les amis d'aujourd'hui ne seront peut-être pas ceux de demain. C'est pragmatique, car les failles techniques ne sont pas toujours les conséquences d'actes de malveillance. Le faux sentiment de sécurité est un écueil majeur en la matière. Le groupe Les Indépendants considère que cette proposition de loi permettra de s'assurer que les dispositifs exploités ne présentent pas de risque pour la sécurité nationale. En revanche, nous tenons à signaler ici notre inquiétude. Si deux équipementiers 5G sont finlandais et suédois, le marché est largement dominé par des acteurs chinois et sud-coréens. La 5G est une révolution comparable à celle du smartphone, tant par ses implications dans nos vies quotidiennes que par les opportunités industrielles qu'elle offre. Nous ne devons pas manquer ce rendez-vous comme nous avons manqué celui du smartphone. Les téléphones sont aujourd'hui sud-coréens ou américains, et leur système d'exploitation est toujours américain. Ne commettons pas l'erreur funeste de croire que le concepteur et l'utilisateur sont sur un pied d'égalité. Il est temps que l'Europe- pourquoi pas sur l'initiative de la France, madame la secrétaire d'État ? -se saisisse de la problématique de la souveraineté numérique. Une commission d'enquête sénatoriale est en cours, et nous nous félicitons qu'elle défriche le sujet. Cette souveraineté nécessitera probablement un volet logiciel et un volet matériel. Où est l'ordinateur grand public français ou européen, le système d'exploitation, ou encore le moteur de recherche ? Nous soutiendrons cette proposition de loi, parce qu'elle sauvegarde les intérêts de la sécurité nationale. Le groupe Les Indépendants enjoint cependant le Gouvernement de définir et de mettre en oeuvre une politique de souveraineté numérique. Cette politique est un enjeu stratégique de long terme, essentiel à l'indépendance de la Nation. La parole Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis quelques mois, le développement de la 5G soulève de nombreuses questions quant à nos exigences en matière de sécurité. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à préserver les intérêts de notre défense et de notre sécurité nationale dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, dans une société où les outils numériques deviennent de plus en plus indispensables au quotidien des Français. En mars dernier, la Commission européenne a recommandé des mesures opérationnelles permettant de garantir un haut niveau de cybersécurité des réseaux 5G sur l'ensemble du territoire de l'Union Elle souhaite que, dès cette année, chaque État membre actualise ses exigences en matière de cybersécurité applicable aux fournisseurs et aux opérateurs, en leur imposant des obligations renforcées, afin de garantir la sécurité des réseaux publics. Comme cela a déjà été dit, ce texte est d'une importance capitale et aura un impact considérable sur le quotidien des Français. Le déploiement de la 5G, prévu en France au début de l'année 2020 et qui permettra de franchir un nouveau cap en termes de connectivité, représente une véritable rupture technologique. En offrant des débits dix fois supérieurs à la 4G, la 5G va accélérer le développement de nouveaux usages, dont les exemples ne manquent pas : développement de la voiture autonome, nouveaux services de télémédecine ou optimisation de la consommation énergétique. Mes chers collègues, le développement de la 5G constitue un enjeu stratégique fort pour la France, que ce soit en termes de compétitivité, de retombées socio-économiques, de protection des données ou encore de souveraineté technologique. Pour relever ces nouveaux défis qui nous attendent, nous devons réunir les conditions nécessaires pour faire en sorte que le déploiement de la 5G se fasse le plus rapidement possible, tout en prévenant les failles d'un nouveau genre dont pourrait faire l'objet le déploiement de nouveaux réseaux. La question de la sécurisation et de la résilience des réseaux de 5G se pose à plusieurs titres. Tout d'abord, les spécificités techniques de la 5G, qui offre une plus grande capillarité des réseaux par la multiplication des antennes et des capteurs, accroissent significativement la vulnérabilité des réseaux. Chaque antenne constitue potentiellement une partie sensible du réseau et n'est pas seulement l'extension passive du coeur de réseau, centralisé et bien protégé, comme c'est le cas pour les réseaux 3G et 4G. Ensuite, l'utilisation de cette nouvelle connectivité dans des secteurs critiques exige une sécurité absolue. L'ensemble de nos installations et établissements porteurs d'infrastructures critiques doivent faire l'objet d'une connectivité irréprochable. Ainsi, on imagine bien les conséquences désastreuses que pourrait avoir la perte de contrôle de plusieurs voitures connectées ou l'interruption d'une opération chirurgicale à distance. Enfin, notre société est tout simplement dépendante de la sécurité des réseaux de télécommunications. je ne vous apprendrai rien en rappelant que les communications électroniques, l'audiovisuel et l'information sont reconnus comme des secteurs d'activité d'importance vitale. L'existence de risques accrus dans les secteurs critiques montre donc la nécessité et l'urgence d'adapter la loi. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a pour ambition de répondre à cette exigence. Je souhaite, à ce titre, remercier et féliciter Mme le rapporteur du travail minutieux qu'elle a réalisé sur ce texte. L'article 1 de la proposition de loi est le coeur de ce texte. En prévoyant un nouveau régime d'autorisation préalable fondé sur des motifs de défense et de sécurité nationale, il vient compléter le dispositif d'autorisation existant, prévu à l'article 226-3 du code pénal, qui encadre la mise sur le marché d'équipements de réseaux de télécommunications, afin de protéger le secret de la correspondance privée. Il soumet à une autorisation du Premier ministre l'exploitation des équipements radioélectriques mobiles permettant de déployer la 5G, sur laquelle transitent les communications électroniques des téléphones portables. L'autorisation sera octroyée pour un ou plusieurs modèles et pour une ou plusieurs versions des appareils connectés, ce qui permettra d'éviter les lourdeurs administratives et de garantir la rapidité du déploiement. Le Premier ministre pourra refuser l'autorisation s'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à la sécurité nationale. Enfin, il disposera d'un pouvoir d'injonction d'injonction en cas d'exploitation sans autorisation. L'article 2 fixe le régime de sanction pénale en cas d'infraction. L'exploitation sans autorisation et le non-respect de l'injonction du Premier ministre seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende L'article 3 prévoit que le régime d'autorisation préalable sera applicable à l'exploitation des appareils installés depuis le 1 février 2019. L'application rétroactive de ce dispositif implique que les opérateurs concernés doivent préparer des dossiers de demande d'autorisation à déposer dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur de la loi pour les équipements déjà mis en place. Enfin, lors de l'examen en commission et par un amendement de Mme le rapporteur, a été adopté visant l'objectif louable de simplifier l'articulation entre les deux régimes d'autorisation que je viens à l'instant d'évoquer, afin d'éviter toute lourdeur administrative. En définitive, qui a été coconstruite en concertation étroite avec les acteurs privés et les autorités de régulation, permet de renforcer et de compléter le cadre juridique, en créant de nouveaux leviers de nature à permettre un contrôle efficace des équipements de réseaux 5G. Aussi, le dispositif demeure suffisamment souple pour ne pas brider les capacités d'innovation des industriels ni retarder l'arrivée de la 5G. Mes chers collègues, je souhaite vivement que les équilibres trouvés sur ce texte et l'état d'esprit consensuel qui a jusqu'à présent animé nos débats

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, dans la course mondiale pour le développement de la 5G, la France doit, elle aussi, avoir un rôle à jouer, pour s'inscrire dans les dynamiques d'avenir. qui dit « nouvelle technologie » dit « nouvelles préoccupations », et celles-ci sont d'ordre varié : économiques, sécuritaires, industrielles, sociales, sanitaires et environnementales. Occulter l'un de ces aspects pour donner la priorité à d'autres, c'est ouvrir la voie à une évolution numérique inadaptée aux besoins de notre temps. Nous déplorons d'ailleurs l'absence d'étude d'impact que la proposition de loi permet confortablement d'éviter, ce dont vous avez parfaitement conscience, madame la secrétaire la sécurité, le texte est insuffisant. Comprenons-le bien, la 5G, avec l'internet des objets et l'interconnexion sans précédent qu'elle promet, nous expose à des vulnérabilités qui exigent plus qu'une autorisation du Premier ministre pour tel ou tel équipement.

Ainsi, les firmes qui seront les heureuses élues pourront acquérir par là même un pouvoir d'influence important, ce qui laisse la voie ouverte aux ingérences étrangères. Ce résultat est la suite logique d'une politique menée depuis plusieurs années ; il est la conséquence directe de l'abandon des outils industriels français de télécommunication, la privatisation de France Télécom et le rachat d'Alcatel-Lucent par Nokia. Aujourd'hui, cela veut dire que les équipements qu'il est crucial de contrôler dans la mise en oeuvre de la 5G ne pourront pas être issus d'une production française, sécurisée par nos standards de défense nationale, et que les éléments sur lesquels repose la sécurisation de nos données devront dépendre d'équipements et d'opérateurs étrangers. La voici, la conséquence des ventes du patrimoine des télécoms français : c'est la dépendance de puissances étrangères sur des points où avancées technologiques et économiques vont de pair avec sécurité nationale. Il faut le rappeler, si les deux géants mondiaux Qualcomm et Huawei remportent la palme d'or en matière de compétitivité, c'est grâce au soutien et à l'intervention de leurs pouvoirs publics. Et nous, que faisons-nous en France, madame la secrétaire d'État ? Notre patrimoine public vendu, il nous reste la timide possibilité d'autoriser ou non l'utilisation de certains équipements. Ce que les agents français de la privatisation et de la vente du patrimoine n'ont pas su anticiper, les puissances étrangères, elles, l'avaient bien compris en témoigne leur position aujourd'hui hégémonique sur le marché de la 5G. Voilà ce qu'il en est des perspectives inquiétantes en matière de sécurité et d'industrie. Mais ce n'est pas tout ; d'autres points méritent notre attention, comme celui de la fracture numérique. Au mois de janvier dernier, Jacques Toubon, Défenseur des droits, soulignait que 13 millions de personnes étaient « éloignées du numérique ». La France à deux vitesses numériques est bien réelle, et, avec elle, les conséquences sociales que cela suscite, alors que les services publics sont dématérialisés à marche forcée. Cette réalité ne cessera de s'aggraver avec la 5G, puisque celle-ci se concentrera, dans un premier temps, Il faut être clair : cet écart de développement continuera d'accentuer une fracture numérique déjà lourde de conséquences. Nous attendons donc que ces enjeux sociaux soient traités au même titre que les enjeux en matière de sécurité, d'industrie, de santé ou d'environnement. L'environnement ? Parce que la 5G promet d'accroître le volume de données transportées, et la dépense en énergie des data centers est déjà chiffrée à 10 % des dépenses mondiales en électricité. Là encore, l'enjeu n'est pas considéré à hauteur de ses implications. Pis encore, un amendement a été adopté le 11 octobre 2018, afin d'alléger la fiscalité applicable aux data centers. S'il est à la mode de brandir le principe du pollueur-payeur, semble-t-il, il en va visiblement tout autrement lorsqu'il s'agit de l'appliquer. Comment la mise en place d'un tarif préférentiel peut-elle encourager les efforts visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Champion de la Terre, je ne sais pas si vous l'êtes, mais champion des lobbies et du business, cela ne fait pas de doute ! Ces questions sont on ne peut plus d'actualité et continueront de l'être toujours plus à mesure que la 5G se développera. Avec elles s'ajouteront également les considérations d'ordre sanitaire, puisque les pollutions électromagnétiques promettent également de s'accroître. Alors que des études estiment que les radiofréquences pour cancérogènes possibles et que nous aurons 1 million d'objets connectés par kilomètre carré d'ici à quinze ans, quelles en seront les conséquences pour notre santé, notre souveraineté et nos libertés individuelles ? Les appels d'offres au plus compétitif sont, eux, déjà sur les rails. Les rencontres entre vous, madame la secrétaire d'État, et les opérateurs privés se multiplient. Mais, sur tous ces enjeux de société, point mort ; rien n'est élaboré. La 5G est prometteuse, mais sa mise en oeuvre exige des précautions qui sont, aujourd'hui, les grandes absentes du projet. Le choix du « tout compétitif » ne saurait répondre à ces besoins, et force est de constater qu'à la souveraineté numérique française vous avez préféré la souveraineté du marché. En vérité, nous devrions avoir un débat de société. Si la 5G et les objets connectés vont nous accompagner dans nos vies, collègue ! ... le marché ne peut tout régler. Nous l'inscrivons dans ce que nous nommons nos « biens communs », notre patrimoine, comme l'énergie, le logement, l'éducation ou la santé. La question est donc de savoir si tout le monde y aura accès,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le déploiement commercial de la 5G est prévu en France pour le début de l'année 2020. Dans un premier temps, il s'agira d'un élargissement de la capacité de la 4G avant la mise en oeuvre des réseaux 5G spécifiques à l'horizon de 2022-2023. Or ce système va entraîner une véritable rupture technologique, avec la mise en place de réseaux virtuels, déconcentrés, gérés par des logiciels et qui entraînent une multitude de flux. Cette virtualisation des réseaux nécessitera moins d'équipements physiques, jusqu'à présent plus facilement contrôlables. revanche, avec plus d'équipements virtuels, des vulnérabilités nouvelles liées à l'architecture de ces réseaux 5G vont apparaître. C'est un changement de paradigme, un changement d'échelle par la rapidité et le débit de la 5G, qui aura pour conséquence de multiples usages nouveaux. Comme avec l'apparition d'internet, il est impossible d'anticiper les applications qui en découleront ainsi que l'ensemble des conséquences de ce nouveau modèle économique. La 5G sera donc le terrain de nombreuses innovations technologiques, et il faudra un grand nombre d'expérimentations et de corrections avant avant que ce système et ce modèle économique ne se stabilisent. Ce facteur d'imprévisibilité se traduira par un accroissement des risques liés. L'objet de cette proposition de loi est bien d'adapter le cadre juridique pour garantir la sécurité du développement et de l'exploitation des réseaux de communications électroniques. Je tiens à féliciter Mme le rapporteur et la commission du travail de clarification du champ d'application de la loi qui a été effectué. On passe en effet d'un dispositif de certification pour assurer une sécurité géographique d'équipements à une sécurisation d'un système par un contrôle de son déploiement et de son exploitation pour des motifs de défense et de sécurité nationale. La commission a bien précisé que les réseaux indépendants n'étaient pas inclus dans le champ d'application de la proposition de loi. On comprend alors que ne sont concernés par cette mesure que les seuls opérateurs de télécommunications déployant des réseaux ouverts au public, sont d'importance vitale, et uniquement pour des motifs sérieux de sécurité nationale. De plus, la commission a fort justement limité ce champ d'application aux équipements 5G et à ceux des générations ultérieures. Cependant, tout en étant d'accord sur le fait que l'État ne puisse pas imposer aux opérateurs une répartition et une pluralité d'équipements sur le territoire national, ni s'immiscer dans leurs politiques d'achat, nous regrettons que la notion de périmètre géographique d'exploitation ait été exclue du dossier de demande d'autorisation par la commission sénatoriale. En effet, il nous paraît important, madame la secrétaire d'État, que l'État puisse connaître le lieu de déploiement et d'exploitation des réseaux 5G. En outre, l'absence d'information pourrait avoir un effet contreproductif et conduire au rejet d'une autorisation qui aurait vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire, ce que nous ne voulons pas. Nous le voyons bien, ce sujet extrêmement complexe méritait mieux qu'un amendement au détour de la loi Pacte. Si l'intention du Gouvernement d'adapter le cadre juridique qui doit garantir la sécurité des réseaux de communications électroniques, en raison des nouveaux usages stratégiques inhérents à la 5G, mérite d'être soutenue, force est de constater que, en recourant à l'initiative parlementaire pour adopter cette loi, il prive le Parlement d'une étude d'impact, qui aurait été éminemment utile pour légiférer sur le sujet. nécessaire d'avoir une évaluation précise des conséquences de ce nouveau dispositif pour les opérateurs et constructeurs réseau. L'avis du Conseil d'État aurait également été important, afin d'anticiper les conséquences en termes de contentieux et de jurisprudence. À l'occasion de l'examen de ce texte, en tant que parlementaires, nous sommes face à une forme d'injonction paradoxale : il faut assurer la sécurité et la fiabilité d'un système, sans pour autant pénaliser l'innovation, le développement de nos entreprises et l'aménagement de tous nos territoires. Dans leur travail, notre groupe et la commission se sont attachés à trouver cet équilibre. Compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques attendues et de l'importance de ce texte, il est également essentiel de disposer d'un cadre juridique évolutif pour garantir dans le temps la sécurité du système. Malgré la qualité des auditions menées, il est difficile de mesurer l'impact du texte sur l'activité de l'ensemble des secteurs concernés ou le déploiement d'une évolution technologique que l'on ne maîtrise pas encore. Une évaluation annuelle du dispositif d'autorisation préalable paraît donc nécessaire. de ces réserves et en prenant en compte les évolutions du texte en séance, le groupe socialiste et républicain, dans une démarche constructive, votera cette proposition de loi.

cette proposition de loi relative à la sécurité des réseaux mobiles, en vue du déploiement de la 5G, est révélatrice des profonds changements en cours, au niveau mondial, dans les rapports de force économiques et commerciaux.

Ne se limitant plus au rôle d'atelier du monde, la Chine a effectué une remontée spectaculaire dans certaines filières comme l'électronique et le numérique, au point d'être en mesure d'y occuper une position dominante et de susciter des craintes plus ou moins fondées. Ce nouveau rapport de force affecte le secteur des télécommunications, avec l'émergence de l'équipementier Huawei et le déclassement d'acteurs historiques comme Alcatel ou Nokia. Dans la course au progrès, des positions qui semblaient pourtant définitivement acquises se voient désormais particulièrement fragilisées. C'est dans un contexte mondial où se mêlent compétition économique et enjeux géopolitiques que nous examinons cette proposition de loi, Comme vous le savez, mes chers collègues, ce texte est inspiré d'un amendement proposé lors de l'examen de la loi Pacte, que la Haute Assemblée avait rejeté. Pour résumer l'enjeu d'une phrase, malgré la technicité du sujet, il s'agit d'apporter une réponse juridique en matière de sécurité au déploiement de la cinquième génération de standards de réseaux mobiles en France. La 5G est bien souvent présentée comme une technologie de rupture, avec des débits de communication étant jusqu'à dix fois plus rapides que ceux et, surtout, de nouvelles applications, comme les véhicules autonomes, la télémédecine ou les infrastructures connectées. Compte tenu de son incroyable potentiel, la 5G fait d'ores et déjà l'objet d'expérimentations et d'investissements importants par les opérateurs, en vue de son déploiement commercial. Afin d'accompagner ce déploiement, en 2017, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Arcep, a lancé un plan de bataille. Si le calendrier est respecté- nous l'espérons, madame la secrétaire d'État -, l'agence devrait procéder à l'attribution des fréquences pas plus tard que cet automne. Si les nouveaux usages que pourrait apporter la 5G pour les consommateurs et les entreprises peuvent être très importants, nous savons aussi quels risques cette technologie pourrait entraîner si elle se déployait en l'absence d'un cadre normatif adapté, notamment en matière de sécurité des réseaux. Prometteuse, cette technologie apparaît aussi plus vulnérable que celles des générations précédentes : risques de piratage, soupçons d'espionnage liés à un fournisseur d'origine étrangère Face à ces incertitudes, le Gouvernement a décidé d'instaurer un nouveau régime d'autorisation préalable, proche de celui qui existe déjà pour les équipements présentant un risque pour le respect de la vie privée et le secret des correspondances électroniques. La réglementation proposée concerne tous les appareils permettant des connexions 5G et « présentant un risque pour l'intégrité, la sécurité, la confidentialité et la continuité de l'exploitation du réseau ». à charge pour eux de récupérer les informations auprès des équipementiers. En pratique, cela confère à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'Anssi, la responsabilité d'instruire les dossiers de demande d'autorisation, en vue d'une autorisation accordée par le Premier ministre dans un délai de deux mois. Notre collègue rapporteur a bien rappelé tout cela, ainsi que la cible, à savoir les opérateurs d'importance vitale. En cas de non-respect de la procédure d'autorisation préalable, l'opérateur se verra appliquer une sanction

On aurait pu imaginer que la charge des démarches ne repose pas sur les seuls opérateurs, mais comment les pouvoirs publics français auraient-ils pu imposer des obligations à des équipementiers implantés, pour la plupart, à l'étranger ? J'ajoute que les conditions d'exploitation relèvent avant tout des opérateurs. Par ailleurs, le danger d'un équipement n'est pas intrinsèque ; il est lié, nous le savons, à la façon dont on l'utilise. Dans son immense sagesse, la commission des affaires économiques a amendé le texte, afin, notamment, de minimiser l'effet des décisions administratives sur le rythme de déploiement et, surtout, de mieux articuler le nouveau régime d'autorisation préalable avec le régime existant, pour éviter les problèmes d'application. Madame le rapporteur, mon groupe vous suit dans cette démarche. Toutefois, je présenterai trois amendements à l'article 1, dont deux portant sur des points qui me semblent plus discutables : la question du périmètre géographique d'exploitation du futur équipement et le problème de la référence aux seuls réseaux 5G pour l'application du dispositif. Mais j'y reviendrai bien sûr lors de l'examen des articles. Enfin, au-delà de ce débat sur la sécurité des réseaux 5G, je profite pour rappeler l'importance de terminer le déploiement de la 4G, voire de générations antérieures, sur l'ensemble du territoire. En effet, à l'heure actuelle, nombre de zones sont encore

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles. C'est en tout cas l'intention qui nous est donnée. La sécurité nationale est en effet un enjeu indéniable, dont la primauté est certaine et que nul ne peut remettre en cause. Ce ne doit être ni un grigri ni un prétexte pour faire passer autre chose. Aussi, il convient de s'assurer que, derrière le principe de ce texte, ne se dissimulent pas d'autres enjeux, moins avouables. Il convient encore de veiller à ce que la sécurité nationale ne soit pas un obstacle au développement ou, plus ironiquement,

qu'un contentieux ne mette à mal son application rapide. Tel était d'ailleurs le sens des propos que j'avais exprimés lors du dépôt de l'amendement tardif au cours des discussions de la loi Pacte. Nous le savons, le déploiement de la 5G est le moteur de la France de demain il permettra de nous placer en pays pionnier de l'innovation et d'agir sur les secteurs essentiels de la santé, de l'agriculture, de la mobilité, des industries et bien d'autres encore, pour l'ensemble de nos territoires, aussi bien ruraux qu'urbains. Se donner les moyens d'un déploiement et d'un développement massif des usages de la 5G revient à asseoir notre position au sein de cette course mondiale, un objectif essentiellement repris dans le cadre de la feuille de route 5G élaborée voilà un an. Je ne puis objectivement nier la nécessité de porter une attention particulière à la sécurité de ces nouveaux réseaux, dont certains usages seront beaucoup plus critiques que ceux que nous connaissons aujourd'hui ; je pense aux véhicules connectés, aux usines connectées et aux interventions chirurgicales qui pourraient être réalisées à distance. Nous avons récemment pu voir à quel point l'espionnage numérique était une réalité tangible au plus haut niveau. Nous avons tout autant pu voir que le piratage informatique n'était pas un problème marginal : c'est ce qu'ont démontré les conclusions des enquêtes américaines sur les manipulations opérées lors des élections présidentielles. Pour reprendre ce dernier exemple, et puisqu'il semble que les Américains ont désigné les Russes comme les coupables très probables, permettez-moi de vous poser cette question : pouvez-vous me citer un équipementier russe qui aurait déployé le moindre matériel dans les réseaux de télécommunication américains ?

alors même que nous ne sommes pas parmi les premiers à déployer la 5G. Si la situation est aussi critique qu'annoncée, notre démarche solitaire me paraît illogique. En dehors des initiatives de certification allemande et du positionnement du Royaume-Uni, dont on peut se demander s'il est libre et éclairé, je ne vois guère d'orientation similaire au sein de l'Europe. S'agissant des solutions proposées dans le texte initial, je n'ai jamais été réellement convaincu de leur efficacité supposée. Je me demande même si le dispositif envisagé aurait simplement pu fonctionner un jour. J'ai en revanche bien identifié les risques attenants à celui-ci, notamment le pouvoir d'autorisation préalable discrétionnaire, qui aurait inévitablement renchéri les coûts de construction et d'exploitation de la 5G, ralenti le rythme de son déploiement. Plus étonnant encore, j'ai relevé les risques avérés sur le bon déroulé du mobile, au point que le comité de concertation du plan France très

Si la proposition de loi a réellement pour objectif de mieux sécuriser nos futurs réseaux de communication électronique, alors l'objectif est atteint. Reste que le texte qui nous est soumis, s'il me semble bien équilibré,

Je m'interroge également sur l'appréciation portée par le Premier ministre sur les modalités de déploiement et d'exploitation des équipements par les opérateurs. Ces critères portent clairement atteinte au principe de libre établissement des réseaux et n'ont, dans ce cadre, aucun lien avec la sécurité nationale.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est, sans en avoir l'air, un texte crucial pour la souveraineté de notre pays. En effet, le fonctionnement et l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles sont sur le point de connaître une véritable révolution, avec le déploiement de la cinquième génération de ces technologies, Loin d'être une simple 4G améliorée, la 5G constitue bien une rupture, dont les effets devraient profondément marquer nos structures économiques, mais aussi notre modèle de sécurité. Bien entendu, la France et l'Europe ne sauraient rester en marge de ce développement. En effet, la 5G est d'ores et déjà en cours de déploiement dans le monde ; certains pays, comme la Chine, sont même parvenus à un stade très avancé. De notre capacité à suivre, voire- soyons ambitieux -à prendre de l'avance dépendront donc notre compétitivité et,, notre place dans le monde. D'un point de vue économique et industriel, la diffusion de cette technologie ouvre de fait la voie à des applications et des usages variés et nouveaux ; l'internet des objets, la domotique, la mobilité ou encore les « villes intelligentes » en sont quelques-uns. Tous ces secteurs d'avenir sont conditionnés à l'accès à la 5G, donc au bon développement des infrastructures adaptées. Néanmoins, au-delà des effets bénéfiques attendus pour la croissance de nouveaux secteurs de notre économie, je souhaiterais m'attarder sur les problématiques que pose l'émergence de cette nouvelle technologie. La commission des affaires étrangères et de la défense à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir ne s'y est pas trompée en se saisissant de la question : la 5G soulève un enjeu important en termes de souveraineté et de sécurité pour notre nation.

La 5G vient en effet renforcer les doutes sur notre capacité à conserver le contrôle des données produites sur notre territoire, et ce d'autant plus que la croissance exponentielle du nombre d'appareils et de systèmes connectés ne fera qu'accroître les risques d'attaques. De plus, et peut-être de manière encore plus inquiétante, ces nouveaux réseaux devraient se révéler particulièrement vulnérables du fait de leur immatérialité et de leur éparpillement. Or ils seront, dans le même temps, encore plus vitaux que les réseaux actuels, et ce à la fois pour nos activités civiles, celles de nos armées et de nos forces de sécurité intérieure. c'est l'un des défis majeurs soulevés par la 5G : notre défense dépendra de plus en plus des réseaux civils de télécommunication. nous accueillons ce texte avec un grand intérêt : il met en place un régime d'autorisation applicable à tous les opérateurs, afin de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Cette proposition de loi institue un nouveau régime d'autorisation administrative, permettant à l'État de maîtriser le déploiement des réseaux 5G et de s'assurer de leur résilience, sans pour autant entraver leur développement. devra néanmoins faire l'objet d'une évaluation, notamment au regard de l'évolution des usages, inconnus aujourd'hui, et du développement des technologies. C'est une garantie de la pérennité de cette protection.

C'est pourquoi il convient de souligner que la France sera précurseur dans ce domaine, qui requiert vigilance et ambition, dans l'attente de décisions des États membres Ce texte, qui reprend un amendement que le Gouvernement avait présenté dans le cadre de la loi Pacte, a fait l'objet d'un important travail des rapporteurs, dont celui de notre collègue Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires économiques. Je voudrais souligner les améliorations apportées à ce texte, qui porte sur un domaine particulièrement sensible en raison des caractéristiques de la technologie concernée, qui ouvre de très nombreuses applications et accentue par conséquent les défauts de sécurisation. La Commission supérieure du numérique et des postes, dont je suis membre, s'était d'ailleurs autosaisie du sujet dans le cadre de l'examen du projet de loi Pacte, car le Gouvernement n'avait pas jugé opportun de solliciter son avis.

sans pour autant que cette évolution se fasse aux dépens des professionnels et de la compétitivité de nos entreprises. En effet, si la cinquième génération de standards de télécommunications mobiles ouvre le champ des possibles pour de nombreuses utilisations, permettez-moi une nouvelle fois de déplorer que bon nombre de territoires, particulièrement en zone rurale, ne soient même pas dotés de la 3G ! Dans mon département des Hautes-Alpes, les maires et les entreprises me font régulièrement part de leur désarroi face à une situation qui empire dans certaines communes. Il est donc impossible d'aborder l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles sans parler des enjeux de cohésion territoriale et des dangers liés au déploiement du très haut débit fixe dans certains territoires, alors que d'autres ne sont pas dotés du moindre équipement. de territoires où il est techniquement compliqué d'apporter des solutions satisfaisantes, et financièrement difficile d'agir pour les collectivités au regard des sommes en jeu. Nous devons veiller à ne pas être pris en otage par les États-Unis et la Chine, qui, eux, sont déjà passés à la vitesse supérieure. Les réseaux 5G mettent en oeuvre une autre technologie, technologie, une technologie de rupture, avec des débits plus importants et un temps de latence bien plus faible qu'aujourd'hui. L'employabilité de la 5G sera donc très étendue et offrira des perspectives très intéressantes, par exemple pour le secteur industriel.

les réseaux de la sécurité nationale, mais aussi pour l'ensemble des équipements, puisque la 5G entraîne un changement d'échelle et multiplie, par conséquent, les risques d'une exploitation malveillante, voire criminelle. Face aux risques encourus, nous devons rester vigilants, sans pour autant pénaliser les opérateurs français, qui ont peu de marges de manoeuvre et qui n'auront pas le monopole de son utilisation. Ce texte doit tendre vers un juste équilibre, qui permette de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, sans retarder le déploiement de la 5G et restreindre ses multiples usages.

Mes chers collègues, vous l'aurez compris, je voterai ce texte. La parole

de simples citoyens sont aussi victimes de hackers. Tout cela sous le règne de la 4G Aussi, faut-il avoir peur de la 5G ou, à tout le moins, doit-on s'en inquiéter ? Cette question est peut-être exagérée, mais on peut se la poser à la lecture de cette proposition de loi et, surtout, à la lecture des arguments et attendus qui l'expliquent et la justifient. la plupart des précédentes interventions soulignent peu ou prou cette inquiétude. Pour confirmer ce sentiment, il suffit de lire la déclaration de la Commission européenne,

reliant des milliards d'objets et de systèmes, y compris dans des secteurs critiques comme l'énergie, les transports, les banques et la santé, ainsi que des systèmes de qui véhiculent des informations sensibles- nous en connaissons tous -et étayent des dispositifs de sécurité ». Je n'oublie pas l'émergence de technologies qui seront sans doute dopées par la 5G : je veux parler de l'industrie 4.0, une nouvelle génération d'usines connectées, robotisées et intelligentes. la Commission européenne insiste encore et invite les États à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour garantir cette sécurité. ma part, je trouve qu'elle le fait de manière péremptoire, mais pourquoi pas ! -« l'obligation renforcée, pour les fournisseurs et les opérateurs, de garantir la sécurité des réseaux. » On ne peut qu'être d'accord La 5G repose et reposera de plus en plus sur des équipements virtuels, des réseaux déconnectés qui accroîtront sa vulnérabilité. Sans entrer dans des détails trop techniques, que d'autres ici maîtrisent d'ailleurs sûrement mieux que moi, il faut constater que, jusqu'à présent, les fonctionnalités reposaient sur des éléments physiques, les logiciels étant eux-mêmes disséminés dans ces équipements. Avec la 5G, les logiciels seront réunis dans le, c'est-à-dire un stockage et un accès par l'intermédiaire d'internet, plutôt que par le disque dur d'un ordinateur, les serveurs pouvant être localisés ailleurs, à des distances importantes ou, du moins, plus importantes. La circulation des données sera de fait beaucoup moins centralisée. Les antennes deviennent elles-mêmes actives et intelligentes. Les informations de plus en plus déconcentrées sont en conséquence davantage vulnérables et peuvent C'est entre autres pour l'une de ces raisons, j'imagine, que la commission des affaires étrangères et de la défense s'est saisie de ce sujet pour avis. La sécurité des réseaux est d'une importance vitale pour notre société et, au premier chef, pour nos forces de sécurité : gendarmerie, police, services de secours et d'incendie et, plus encore, armées. Ces forces interviennent et s'appuient sur les réseaux civils de télécommunication pour leurs activités opérationnelles sur le territoire national. Elles sont donc directement concernées par le développement de la 5G et tout particulièrement sensibilisées à sa potentielle vulnérabilité. Des expérimentations de la technologie 5G ont été lancées en France en 2018. Comme vous le savez, l'attribution des bandes de fréquences est prévue pour la fin de l'année.

Le sujet, madame la secrétaire d'État, méritait manifestement mieux qu'un amendement. Avons-nous pour autant satisfait ou épuisé le sujet, tout en ayant répondu à toutes les interrogations ? Certainement pas Le directeur de l'Anssi disait lui-même que toutes les ressources de la 5G n'avaient pas été explorées et qu'il s'en fallait de beaucoup. Pour autant, ce texte que l'on nous demande d'adopter dans l'urgence est indispensable. On peut regretter cette urgence, qui nous a privés d'un travail parlementaire beaucoup plus approfondi- certains orateurs l'ont déjà dit -, mais ce texte est une réponse appropriée pour le moment. Je rejoins ma collègue Viviane Artigalas pour souhaiter un suivi permanent de cette technologie, par essence particulièrement évolutive et nécessitant en conséquence des adaptations régulières. Il faut J'en termine, monsieur le président. La 5G sera une véritable rupture technologique, ouvrant des champs d'application considérables. Elle est une chance que nous devrons saisir et nous approprier, tout en prenant toutes les mesures possibles

qui rendront ceux plus vulnérables. Cette vulnérabilité concerne la sécurité des biens et des personnes, mais aussi la continuité de l'action de l'État. Ici, il est essentiellement question des réseaux régaliens de la sécurité intérieure et civile. Or, dans la course au déploiement de la 5G, plusieurs études soulignent que les opérateurs dits « verticaux » sont aussi dans les starting-blocks, et qu'il y aura un développement et une multiplication de réseaux privés. En effet, la 5G, ce sera du très haut débit en mobilité nationale, mais aussi au en bande étroite, dans les aéroports, les gares et les sites industriels, avec la possibilité de remplacer très avantageusement le WiFi pour les objets connectés, les véhicules autonomes et divers services que l'on n'imagine même pas aujourd'hui. même pas aujourd'hui. Comme les débats à l'Assemblée nationale l'ont montré, si l'on peut estimer que les risques pesant sur les réseaux privés ne présentent pas le même caractère systémique que ceux qui pèsent sur les opérateurs de télécommunication, la 5G modifiera très certainement les équilibres actuels. Ce dernier point mérite une attention particulière dans un contexte de privatisation de nombreuses entreprises en réseau. Nous pensons en particulier à EDF, dont le futur est très incertain puisque l'on parle d'une scission possible de l'entreprise, avec une privatisation partielle ; nous pensons à la SNCF dont la privatisation larvée est en cours ; nous pensons aussi à ADP- quoique vous soyez bien mal partis qui, sans être une entreprise en réseau, peut potentiellement développer un réseau vertical. C'est aussi le cas des sociétés d'autoroutes, qui lorgnent aujourd'hui le réseau des routes nationales, et des industriels de l'automobile. À cet égard, la SNCF a préconisé un modèle d'opérateur virtuel constitué au sein de la société d'économie mixte Synerail, qui réunit SFR, TDF et Vinci pour gérer son réseau mobile. Vous comprendrez que les annonces des privatisations de ces entreprises nous laissent encore plus dubitatifs, tant les enjeux stratégiques liés à ces entreprises semblent toujours plus importants. En effet, ces sociétés sont très sensibles aux aspects de sécurité, qu'il s'agisse d'aéroports ou d'alimentation électrique. De plus, ces opérateurs, nous avons eu l'occasion de le rappeler lors du débat sut la privatisation d'ADP, sont souvent en situation de monopole ou de quasi-monopole. La parole

Cette déclaration a été faite par le département du commerce américain, non pas de l'administration Trump, mais de l'administration Obama. C'était il y a huit ans déjà.

-, afin de mieux assurer la sécurité des flux de ses clients. Le régime chinois, qui affirme vouloir dominer le monde d'ici à 2050 et qui dispose désormais d'un président potentiellement à vie, ne reconnaît pas la démocratie et les droits de l'homme comme valeur universelle. Définie par sa Constitution comme un « État socialiste de dictature démocratique populaire », la Chine compte plusieurs dizaines de milliers de prisonniers politiques et un millier de musulmans détenus dans des camps au Xinjiang. Sa maîtrise de la technologie lui a permis de créer un « cybermur » pour imposer un contrôle social à sa population, en combinant réseaux sociaux, caméras à reconnaissance faciale et intelligence artificielle. Cette dictature 5G utilise ses « routes de la soie » pour tenter de prendre subrepticement le contrôle de pays en liant son aide à la signature de contrats d'équipements technologiques. Après Djibouti, la Chine aura installé 10 000 caméras sur l'île Maurice d'ici à la fin mois de janvier, j'ai interrogé le ministre des affaires étrangères sur la position de la France vis-à-vis de Huawei, en particulier en ce qui concerne le déploiement de la 5G. Il avait alors partagé sa préoccupation avec notre commission.

voté, partageant le sentiment d'urgence qui animait le Gouvernement pour bloquer l'implantation d'équipements qui auraient pu contrevenir à la défense de nos libertés publiques. Je me réjouis que le Gouvernement ait persisté en nous proposant ce texte, même si je regrette qu'il ne bannisse pas officiellement Huawei,

En effet, pour la pleine efficacité du dispositif prévu, les équipementiers sont les plus à même de répondre à l'ensemble des sollicitations sur l'appareil ou le logiciel visé. Quel est l'avis de la commission

couvert par les dispositions de l'article 1. La commission a restreint le champ d'application du dispositif de demande d'autorisation préalable en faisant explicitement référence aux réseaux 5G et aux éventuelles générations ultérieures. Or, dans la perspective du déploiement, les opérateurs de télécommunications mobiles s'appuient plutôt sur une transition d'une technologie vers l'autre sans interruption, bien qu'il s'agisse effectivement de technologies distinctes. Dans tous les cas, il ne semble pas opportun de fixer ce genre de disposition dans la loi, car il s'agit avant tout d'une question technique devant être réglée par des techniciens., cela complique le texte. C'est pourquoi il est proposé ici de supprimer la mention de la 5G et des générations ultérieures. Quel est

Mme Maryse Carrère. Le triptyque « intégrité-confidentialité-disponibilité » constitue le socle fondamental utilisé par tous les acteurs de la cybersécurité. À l'article 1, deux de ces termes sont mentionnés parmi les objectifs de l'autorisation d'exploitation de réseaux de réseaux 5G à la suite de l'intégration par la commission de la notion de confidentialité. Nous proposons de mentionner également la disponibilité du réseau. En effet, l'accès à l'infrastructure de réseau est un élément fondamental

introduisons pour les opérateurs concernés par ce texte une obligation de notification au Premier ministre de toute modification apportée à leur matériel par les équipementiers. Si les modalités de cette modification sont fixées par décret, on peut supposer que le Gouvernement ne fera pas peser sur les opérateurs une trop lourde charge et s'en tiendra à l'envoi d'une détaillée, qui suffira amplement.

L'objet de cet amendement, mes chers collègues, est donc de pallier la difficulté posée par la modification contenue des logiciels par un système d'autorisation préalable. Cette solution n'est pas incompatible avec la proposition d'établir un rapport annuel sur les autorisations délivrées. Elle est même complémentaire, puisque l'adoption de cet amendement offrirait à l'administration la matière pour constituer une formidable base de données des équipements 5G utilisés par les opérateurs d'importance vitale et de leurs différentes versions. Quel

De plus, il est proposé que le Premier ministre puisse abroger sa décision sur le fondement d'une simple déclaration. Or, si la modification effectuée venait à mettre l'opérateur en situation de manquement aux conditions qui lui étaient imposées par l'autorisation, il serait quoi qu'il

Nous sommes effectivement favorables à ce qu'il soit fait référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux 5G pour définir la liste des appareils dont l'exploitation sera soumise à autorisation préalable.

présenter l'amendement n° 9 rectifié. La commission, sur proposition de Mme le rapporteur, a supprimé la référence au périmètre géographique dans le dossier de demande d'autorisation, considérant que cette information ne devait en aucun cas permettre à l'État de s'immiscer dans la politique d'achat des opérateurs. pour dire qu'il ne faut pas que, à terme, l'application du régime d'autorisation préalable permette à l'État d'imposer aux opérateurs le choix des équipementiers par zone géographique. Mais si nous approuvons cet objectif, il nous semble cependant que la suppression, au stade de l'instruction du dossier, de l'information relative au périmètre géographique d'exploitation n'est pas la bonne solution. En effet, comment instruire une demande d'autorisation sans connaître le lieu géographique du déploiement et de l'exploitation du réseau ? Il est bien évident que la décision du Premier ministre d'autoriser, ou non, l'exploitation d'un réseau sera en partie guidée par la présence, ou non, de sites ou d'installations sensibles. Si les services de l'État ne disposent pas de cette information, cela pourrait les conduire au rejet d'une demande qui aurait vocation à s'appliquer sur tout le territoire. Or un large consensus s'est exprimé dans le cadre de cette proposition de loi pour, justement, éviter l'exclusion totale d'un équipementier. Aussi, au travers de notre amendement, nous proposons d'en revenir au texte de l'Assemblée nationale, qui prévoit que le dossier de demande d'autorisation remis par l'opérateur

commission, qui a supprimé la référence au périmètre géographique en réponse à l'inquiétude des opérateurs, qui craignent, à juste titre, que l'État ne leur dicte leur politique d'achat.

comment fera l'État pour savoir où vont se déployer les réseaux de la 5G si ce n'est pas indiqué dans le dossier ?

Rattaché au service de l'économie numérique à Bercy, ce commissariat a acquis en décembre 2017 une compétence nationale qui lui confie la responsabilité de l'ensemble des obligations légales des opérateurs. À ce titre, il a notamment pour fonction de s'assurer que les équipementiers et les opérateurs mettent en place les systèmes d'interception et les équipements nécessaires aux techniques de renseignement. Il est également chargé de définir et de faire réaliser des systèmes permettant d'assurer les interceptions légales de communications sur les réseaux des opérateurs, qu'il s'agisse d'interceptions requises par des magistrats ou d'interceptions de sécurité entrant dans le cadre de la protection de l'État

assurer en situation de crise la coordination de l'action des différents opérateurs, afin que ceux-ci fournissent des prestations adaptées aux besoins des services ministériels, des entreprises ou des organismes placés sous tutelle et informer les autorités gouvernementales sur l'état des liaisons nationales et internationales de communications électroniques. Son rôle dans le dispositif serait d'autant plus important si l'on en croit les conclusions du rapport que le coordinateur européen de lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, a remis au Conseil le 7 juin dernier. Ce rapport souligne en effet les incidences de la mise en place de la 5G sur les autorités judiciaires et les forces de l'ordre, en particulier pour ce qui concerne l'interception légale de communications et l'urgence des mesures à prendre afin que cette capacité soit préservée. Le rapport identifie trois risques liés au développement de la 5G : le chiffrage des communications de bout en bout, celui de la carte SIM et l'architecture virtuelle et fragmentée de la 5G. Le coordinateur européen recommande ainsi de tenir compte des éléments suivants l'enregistrement de tous les fournisseurs et l'obligation qui leur est faite d'extraire une copie de surveillance complète et non cryptée ; l'obligation de structurer leur réseau de manière que les données de localisation soient toujours disponibles ; enfin, l'obligation de coopérer, afin de permettre des mesures techniques comme l'identification du numéro de carte SIM. La mise en oeuvre La mise en oeuvre de ces recommandations entre, à l'évidence, dans le cadre du rôle dévolu au commissariat. Vous l'aurez compris, tant de compétences et de fonctions en font un acteur tout désigné dans le processus d'examen des dossiers pour l'octroi d'une autorisation préalable.

dans tout ce qui a trait à la gestion des interceptions. Je puis vous confirmer la pleine implication du CCED dans la mise en oeuvre de la feuille de route 5G, notamment sur la question des interceptions légales. Néanmoins- et c'est pour cette

il n'est pas incongru que la représentation nationale, à l'occasion de cette discussion, mette l'accent sur ce point par le biais de cet amendement. Personnellement, je le voterai. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

d'enquête présidée par notre collègue Franck Montaugé, et ce que nous y entendons est absolument terrifiant. On pourrait parfaitement imaginer qu'une puissance étrangère prenne le contrôle à distance d'un hôpital et fasse subir aux patients des surdoses de rayonnement X au moyen de ces ces objets connectés. Il nous faut vraiment prendre conscience de notre vulnérabilité à ces nouvelles technologies, et je regrette que ce texte ne porte que sur un aspect extrêmement limité de la problématique.

les auditions que nous avons menées n'ont pas permis de démontrer l'intérêt et l'efficacité d'une pluralité d'équipements dans un même périmètre, en l'absence notamment d'interopérabilité

Cet amendement a pour objet de supprimer les critères liés aux modalités de déploiement et d'exploitation retenues par l'opérateur. En effet, il apparaît disproportionné, sous prétexte de vérifier la conformité d'équipements aux objectifs de sécurité fixés par l'État, de mettre sous tutelle les modalités d'exploitation et de déploiement des réseaux mobiles. Le recours à ces critères porterait atteinte, non seulement à la liberté du commerce et de l'industrie, dont découle le principe de libre établissement des réseaux, mais aussi à la libre circulation des marchandises et des services.

de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service. Elles précisent également que l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Dès lors, les dispositions envisagées seraient disproportionnées

Selon le Gouvernement, l'analyse du Premier ministre portera en particulier sur les opérations de configuration et de supervision réalisées sur les appareils soumis au contrôle et sur les sous-traitants impliqués dans ces opérations. Les modalités de déploiement concerneraient la conception des réseaux, avant leur activation. Elles conduiraient l'Anssi à vérifier, notamment, la bonne activation des options de sécurité, l'existence d'une architecture limitant l'exposition aux attaques, la mise en place d'une redondance ou encore de protections périmétriques. La mention de « modalités d'exploitation » renverrait aux actions des opérateurs sur les réseaux, une fois ces derniers activés. L'Anssi pourrait ainsi s'assurer du caractère sécurisé de l'administration du réseau, des modalités de contrôle

Dans un tel contexte, nous persistons à penser que le risque d'ingérence ne doit être explicitement mentionné que pour les États hors de l'Union européenne.

La commissaire européenne Mariya Gabriel l'a récemment rappelé : protéger les réseaux 5G, c'est protéger l'infrastructure qui soutient diverses fonctions sociétales et économiques vitales telles que l'énergie, les transports, les activités bancaires et le secteur de la santé, sans compter les usines du futur. Dans cet hémicycle, nous avons été nombreux à dresser le même constat. C'est également protéger nos processus contre les ingérences et la propagation de la désinformation. C'est la raison pour laquelle nous considérons que, en cas de risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la France, l'exigence de proportionnalité n'a pas lieu

Un certain nombre de garanties ont été ajoutées en ce sens au cours de l'examen parlementaire du présent texte, afin de minimiser et d'encadrer les effets de cette nouvelle procédure sur les déploiements des opérateurs. Je pense notamment à la fixation de délais

L'alinéa 12, tel qu'il est issu du travail de la commission, nous paraît trop prescriptif : il conditionne tout refus éventuel à une absence de disproportion entre, d'une part, le coût et le rythme de déploiement du réseau et, d'autre part, l'atteinte à la défense et à la sécurité nationales. Cette proposition de but de protéger la défense et la sécurité nationales. On ne peut relativiser ce motif impérieux d'intérêt général par des considérations liées au déploiement des réseaux sans remettre en cause la portée même de ce régime d'autorisation et son maniement par le Premier ministre, qui prendra en compte tous les éléments pertinents pour assurer la proportionnalité de sa décision, comme de toute décision administrative.

du déploiement des appareils sur le territoire national, le renchérissement des coûts de ce déploiement et la remise en cause de l'accès des utilisateurs finaux au service qui en résulterait sont proportionnés aux risques sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales.

en matière de communications mobiles, avec la mise en place de véritables réseaux virtuels régis par des logiciels, organisant une multitude de flux et dont les fonctions intelligentes seront déconcentrées.

Il est difficile, malgré toutes les auditions qui ont pu être menées, d'en mesurer l'impact, aussi bien sur l'activité des acteurs concernés que sur le déploiement de la 4G, qui doit se poursuivre sur l'ensemble du territoire, et sur les premières expérimentations de la 5G. Il est également difficile d'appréhender les nouveaux usages qui vont en découler. La 5G sera le terreau de nombreuses innovations technologiques et un grand nombre d'expérimentations et de corrections seront nécessaires avant que le réseau ne se stabilise. Ce facteur d'imprévisibilité induira un accroissement des risques lié à l'utilisation de technologies non parfaitement matures et au fait que la protection contre ces risques nécessitera des ajustements. Il est donc essentiel, compte tenu de l'importance de ce texte et de la rapidité des évolutions technologiques liées au développement de la 5G et à ses potentiels, de pouvoir disposer d'une évaluation régulière. Celle-ci permettrait, si besoin, d'adapter le cadre juridique pour remédier aux vulnérabilités nouvelles identifiées et garantir la pérennité des protections déjà mises en places. Une évaluation annuelle du dispositif d'autorisation préalable paraît donc nécessaire. Aussi est-il proposé que le Gouvernement présente chaque année, à compter de juillet 2020, un rapport analysant l'impact de la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi ainsi que ses éventuelles incidences

Nous eussions aimé que vous nous présentassiez votre projet politique pour la constitution d'une

J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à préserver les intérêts Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale

tendant à insérer un article additionnel après l'article 20.

la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative aux modalités de prononcé des sanctions à l'encontre des personnels de surveillance grévistes, sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'administration pénitentiaire est soumise à un statut spécial qui interdit le droit de grève afin d'assurer la continuité du service public et la sécurité de nos établissements pénitentiaires. Il importe, dès lors, que des mouvements concertés d'arrêt de travail

Le Conseil constitutionnel ne l'a d'ailleurs pas exclu de sa décision. À ce titre, nous sommes donc plutôt en accord avec la non-consultation du conseil de discipline proposée par le Gouvernement.

que tout agent mis en cause a le droit à la communication de son dossier, du moins aux pièces concernant les faits qui lui sont reprochés. Il s'agit d'un élément essentiel pour lui permettre de préparer sa défense. Nous sommes conscients qu'un décret viendra préciser la procédure applicable, mais nous souhaiterions, monsieur le secrétaire d'État, que vous nous apportiez des précisions sur ce point et, le cas échéant, des assurances sur le contenu du futur décret d'application. Dans cette attente, la commission a rendu un avis de sagesse plutôt positive sur cet amendement.

Le maire de Paris dispose d'une compétence de police municipale, comme tous les maires, mais la sienne présente deux spécificités : la première est que ces pouvoirs sont consentis au gré de la loi,

sur la procédure disciplinaire applicable aux surveillants de prison en cas de violation de l'interdiction légale de la grève dans les prisons est un amendement statutaire. Il s'intègre parfaitement à un texte qui comporte, d'ailleurs, d'autres dispositions en matière de discipline. En revanche, l'amendement qui a été déclaré irrecevable n'était

pour mieux intégrer les agents contractuels dans le cadre normatif applicable aux agents publics, le présent amendement vise, par cohérence, à renommer le futur code : « code de la fonction publique et des

d'un amendement de coordination avec la création proposée d'une catégorie A+ dans la fonction publique. Le futur code général de la fonction publique devra prendre en compte la création de cette nouvelle catégorie et procéder au toilettage nécessaire du statut.

la création d'un code général de la fonction publique. Elle a retiré du champ de cette habilitation la suppression de dispositions législatives que le Gouvernement jugerait inadaptées. En effet, cette démarche relève d'un choix d'opportunité, qui appartient par principe au seul législateur et ne saurait être délégué à cette occasion. Nous avons également supprimé la demande de dérogation au principe de la codification à droit constant. Il s'agit en réalité d'une demande d'habilitation à légiférer par ordonnance détachable de toute démarche de codification.

avant l'examen du projet de budget. Il ne paraît pas opportun d'alourdir encore le fonctionnement des assemblées locales. Imposer la tenue chaque année d'un débat sur ce sujet n'aurait pas vraiment d'intérêt. De plus, cet amendement semble

Il serait d'ailleurs difficile, dans une commune de plus de 3 500 habitants employant moins de cinquante agents, d'organiser une concertation préalable au sein du comité social territorial, puisqu'un tel comité n'existe pas- il est placé auprès du centre de gestion. La commission est donc défavorable

prévoit déjà que le rapport fourni à l'occasion du débat d'orientation budgétaire intègre un certain nombre de dispositions relatives au personnel, à la masse salariale et à la gestion

Actuellement, la loi encadre le droit de grève dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique hospitalière, mais rien n'est prévu pour la fonction publique territoriale. L'objet de cet amendement est de combler cette lacune.

a fait l'objet de toutes les consultations et de toutes les expertises juridiques nécessaires. Il me semble répondre à la problématique des collectivités territoriales, finalement très simple : il s'agit non pas d'empêcher la grève,

se déclarent en grève à onze heures trente, sans plus de considération pour les enfants, et que ce sont des gens peu qualifiés, voire des élus, qui, bénévolement, viennent servir à la cantine. Tout cela n'est pas sérieux : il faut prendre en compte la réalité et la qualité du service public,

Trois outils distincts sont prévus : le préavis de grève, la cessation du travail dès la reprise de service- ce qui s'applique à la Ville de Paris -et une durée minimale de cessation du travail pour éviter les grèves perlées.

recherché et répondre à la nécessité de définir les services concernés en renvoyant à l'autorité territoriale le soin de le faire dans une négociation. Cet amendement est plus favorable à la concertation avec les partenaires sociaux et ne nous semble pas entaché d'un risque

périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la délivrance des titres d'état civil. Comme à chaque fois, nous vous opposons la réalité : museler les agents du service public ne fera pas disparaître les causes

aux articles 1 à 5, voici que vous vous attaquez au droit de grève des agents de la fonction publique territoriale, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels.

et de la liste des activités qui seraient concernées. Ce qui aujourd'hui désorganise le service public local, ce ne sont pas les agents lorsqu'ils font valoir légitimement leur droit à revendication,

Si permettre aux agents d'une collectivité territoriale de définir eux-mêmes, avec l'autorité territoriale, les conditions d'exercice de leur droit de grève pour que les choses se passent bien et permettre

tombe bien : vous l'êtes ! Comment peut-on aujourd'hui défendre à tout prix un concept qui ne permet pas l'exercice du droit de grève dans de bonnes conditions ? un concept qui ne permet l'exercice du droit de grève qu'au détriment de ceux qui bénéficient des services publics, en les privant de la continuité du service public ? Vous ne savez pas ce que

c'est parce que, outre ce qui se pratique généralement dans l'administration parisienne, il prévoit la possibilité, pour l'autorité territoriale, de mener une négociation, donc de travailler avec les partenaires sociaux. La parole est à M.

à assurer l'homogénéité des règles applicables aux trois fonctions publiques en cas de grève. Il n'y a pas de quoi tenir un débat de principe ou idéologique sur ce sujet.

En ce moment précis, je pense aux nombreuses luttes ouvrières des siècles passés.

qui savent s'accorder sur des objectifs de destruction de droits acquis.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

Leur personnel relève aujourd'hui de la fonction publique hospitalière, alors même que ces services sont rattachés aux départements ou, depuis la loi Maptam, à la métropole de Lyon. Cette situation soulève deux difficultés. Tout d'abord, elle complique sérieusement la mobilité des agents, les équivalences entre les corps de la fonction publique hospitalière et les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale étant difficiles à établir. Ensuite, elle complexifie la gestion des ressources humaines. Ces difficultés sont notamment rencontrées par l'Institut départemental de l'enfance et de la famille, l'IDEF, un service de l'IDEF, un service de la métropole de Lyon qui comprend 353 agents, chargés principalement de l'accueil d'urgence des jeunes âgés de moins de 18 ans et des mineurs non accompagnés.

les personnels de certains services sociaux, comme l'Institut départemental de l'enfance et de la famille, sont régis par le statut de la fonction publique hospitalière, alors qu'ils sont employés par le département ou la métropole de Lyon. Cette situation nuit grandement à la mobilité des agents à l'intérieur du département ou de la métropole de Lyon : il faut trouver, pour chaque mobilité, des cadres d'emploi équivalents dans la fonction publique territoriale, ce qui n'est pas toujours simple.

Le scrutin est ouvert.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

Ce système dual est source de lourdeurs administratives, notamment en matière de dialogue social, et freine la mobilité des agents. Il est proposé d'appliquer le statut de la fonction publique territoriale à l'ensemble des agents du CASVP. le législateur a déjà adopté cette disposition en 2016 sur l'initiative de M. Dussopt, alors député. L'amendement comportait toutefois une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier.